nous voici réunis pour débattre d'une proposition de loi dont l'objectif est de créer les conditions nécessaires à la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste.

en particulier qu'il soit porté atteinte à la représentation des salariés. Nous ne sommes pas beaucoup trompés ! Notre pays souffre d'une dégradation générale du dialogue social, ainsi que d'un manque de lien, d'une perte de proximité entre les IRP et les salariés qu'elles et les salariés qu'elles représentent. Force est de constater, dans le même temps, que les questions de santé et de sécurité au travail passent très souvent au second plan, avec la disparition des CHSCT. On ne peut pas dire que les choses aillent dans le bon sens. Depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, les entreprises ont regroupé leurs instances- dont les CHSCT -au sein de CSE. Dans la fonction publique, la loi du 6 août 2019 a substitué les comités sociaux aux a substitué les comités sociaux aux comités techniques. Nous sommes donc contraints de légiférer, mais pas n'importe comment, car La Poste n'est pas n'importe quelle entreprise. Dans les faits, elle est atypique, puisqu'elle est devenue en 2010 une société anonyme tout en continuant à accomplir des missions de service public et d'intérêt général très importantes

qui sont le fruit de l'histoire et de la singularité de cette entreprise. Lors de nos récentes auditions, nous avons compris que le projet de la direction de l'entreprise, présenté aux organisations syndicales le mois dernier, prévoit de passer de 145 comités techniques à 28 CSE

La Poste, c'est une forte diversité de métiers, répartis sur des sites multiples. Ce qui se prépare est la réforme la plus importante à ce jour d'instances représentatives du personnel d'une entreprise dans le cadre des ordonnances de 2017. de cette entreprise ont vocation à couvrir l'ensemble des territoires métropolitains et ultramarins, six jours sur sept. Ce n'est pas rien ! Les sénateurs que nous sommes, tous attachés à leur département, ne doivent pas considérer le vote de cette proposition de loi comme une simple formalité. Il ne faudrait pas, par exemple, que la mise en place de ces CSE

En pratique, il y aurait de nouvelles suppressions de postes, qui se traduiraient inévitablement par la fermeture de bureaux de poste et de points de contact, et par une accélération de la désertification postale que nous constatons sur nos territoires.

pour une bonne représentation des salariés, sera mise à mal. J'ai une pensée toute particulière pour les territoires ultramarins, dont l'éloignement et les spécificités sont totalement ignorés à ce stade. stade. Par voie d'amendement, nous proposons d'envisager la mise en place d'un droit syndical de transition durant la première mandature des CSE. C'est un sujet important, en particulier parce que plus de 1 000 représentants syndicaux vont voir leur détachement prendre fin à la date de mise en place des CSE.

à un effondrement de l'offre sociale, accru par de possibles disparités entre CSE. Nous avons déposé quelques amendements pour améliorer ce texte et poser les bases de discussions futures entre la direction de La Poste et les représentants actuels du personnel.

la proposition de loi du groupe Union Centriste visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste a pour objectif de procéder à la réforme des institutions représentatives du personnel de cette

représentatives du personnel spécifiques, qui sont le résultat de l'histoire de l'entreprise et de la prise en compte des spécificités de ses missions. On y observe notamment une forte proximité des instances avec le personnel.

qui a entraîné la transformation du service public postal en société anonyme à capitaux publics et, par conséquent, provoqué la coexistence de fonctionnaires, de salariés de droit privé et de contractuels de droit public. Cette diversité de personnel a entraîné la création d'institutions représentatives du personnel spécifiques à La Poste. L'application aveugle des ordonnances de 2017 à La Poste va diviser par trois le nombre d'instances sociales et réduire les prérogatives des délégués du personnel.

Cet éloignement des représentants syndicaux de proximité néglige l'enjeu de prévention des risques professionnels, alors que La Poste est l'entreprise publique qui a connu le plus grand nombre de suppressions d'emplois : 146 175 emplois disparus en vingt ans ! Le personnel subit des conditions de travail dégradées, l'explosion du recours à la sous-traitance et des réformes à marche forcée ; dès lors, la prévention des risques professionnels devrait être la priorité de la transformation des instances de représentation

identiques ». Le remplacement des CHSCT par des CSSCT réduira les prérogatives des représentants du personnel, qui ne disposeront qui ne disposeront plus de la capacité de réaliser des expertises et d'ester en justice. La situation sociale à La Poste, avec la perte de milliers d'emplois par an et une restructuration une restructuration permanente, nécessite la préservation d'instances de proximité et le maintien des CHSCT. Nous refusons de cautionner une organisation dont les experts experts pointent les risques pour la santé des salariés. Notre groupe est profondément attaché à La Poste. Malgré les choix stratégiques de la direction de généraliser la sous-traitance et l'ubérisation, le premier employeur de France après l'État, avec 210 000 agents qui accomplissent une mission de service public sur l'ensemble du territoire national. Nous participons au quotidien aux luttes menées pour maintenir ouverts les bureaux de poste dans nos communes, car nous sommes convaincus de l'importance du service public. Nous voterons donc contre votre proposition de loi. La parole

de loi, Denise Saint-Pé, pour sa juste intuition. Le 1 janvier 2023, une page de l'histoire de La Poste se tournera, avec la fin du célèbre timbre rouge, dont l'existence remonte à 1849. Sans cultiver la nostalgie, mes chers collègues, reconnaissons que le timbre rouge et la voiture jaune de La Poste, tout comme la voiture bleue d'EDF, c'est la France la France qu'on chérit et qu'on aime ! Ce timbre rouge laissera la place à un code à huit caractères, que les utilisateurs devront télécharger en ligne avant de le recopier sur leur enveloppe. Certains y verront une anecdote ; d'autres, comme moi, un exemple d'une mutation qui bouleverse et met fin, peu à peu, aux codes d'une institution qui nous a précédés et qui, je l'espère, nous survivra. Pour cela, mes chers collègues, nous devons nous saisir de la question sociale, en favorisant toujours la préservation d'un dialogue vivant et renforcé, si fondamental pour les salariés et dont l'intérêt dans le contexte que nous vivons actuellement n'est plus à souligner. De manière plus globale, je veux vous faire partager mon inquiétude sur les bouleversements

L'entreprise se transforme et accélère la diversification de ses activités au détriment, parfois, d'une ruralité où le sentiment d'abandon est de plus en plus fort. Or les Français demeurent très attachés à La Poste. Cette entreprise est, pour chacun de nous, le symbole du dynamisme local. À l'inverse,

Dans ce contexte difficile, c'est avec une volonté affirmée que le groupe Union Centriste soutiendra cette proposition de loi, qui exprime les valeurs que nous partageons, notamment par la confiance accorde aux partenaires sociaux et par leur valorisation au sein du monde de l'entreprise. Ce texte a pour but de rendre applicables à l'ensemble du personnel de La Poste les dispositions du code du travail

sociale et même au solidarisme ! Très bien ! Les entreprises sont utiles pour produire de la richesse, bien sûr, mais elles ont une responsabilité sociale et environnementale. Il est donc essentiel de pérenniser le dialogue entre les salariés, les partenaires sociaux et le patronat. On ne peut espérer l'amélioration d'un système sans passer par la concertation et, plus encore, la négociation- c'est ce qu'on peut appeler le modèle rhénan. Il m'apparaît également essentiel, dans un souci d'égalité, que le cadre légal de la représentation syndicale dans une société anonyme comme La Poste ne diffère pas de celui qui est applicable aux autres sociétés anonymes, même lorsqu'une petite partie des collaborateurs est sous contrat public, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous ne doutons pas que, dans une entreprise au dialogue social riche et nourri, les intéressés sauront transiter du droit d'exception au droit commun, en veillant à ce que cela se fasse au bénéfice de chacun. C'est du moins ce que nous attendons toujours du paritarisme. La transformation du paysage des IRP va donc dans le bon sens. Nous sommes conscients que la mise en place de CSE à La Poste constitue un chantier de grande ampleur, qui engage un changement structurel majeur, avec le passage au droit syndical applicable aux entreprises privées. Les partenaires sociaux doivent être en mesure de négocier la mise en place d'un cadre de dialogue social ambitieux, prenant notamment en compte le défi de la proximité et les besoins de nos territoires, en particulier dans les outre-mer. Les salariés de droit privé représentent aujourd'hui plus des deux tiers des quelque 170 000 collaborateurs de La Poste. Plutôt que d'avancer à marche forcée, ce texte donne du temps

n'est pas sans nostalgie pour les années que j'ai passées au sein de cette grande maison qu'est La Poste que je m'exprime aujourd'hui au nom du groupe RDSE. L'exercice d'un métier dans l'une des innombrables activités du groupe La Poste est une expérience qui apporte de la rigueur, fait naître des rencontres et procure un sens aigu du service public.

tant il conditionne le climat social en son sein, ce qui nous amène au sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'évolution des institutions représentatives du personnel à La Poste. L'ouverture de ce chantier devenait urgente, au vu de l'impossibilité pour l'entreprise de bâtir un modèle de dialogue social fondé sur les dispositions du code du travail en matière de comités sociaux et économiques ou sur celles du code général de la fonction publique relatives aux comités sociaux d'administration. du personnel fait en effet que ceux-ci relèvent tantôt du droit privé, tantôt du droit public- résultat d'une succession de lois ayant complexifié le modèle pour répondre aux injonctions du néo-libéralisme et aux impératifs de rentabilité dans un marché concurrentiel. Après avoir exposé ce problème, insoluble avec la législation en vigueur, notre collègue Denise Saint-Pé s'est saisie de ce sujet avec justesse pour garantir la continuité durable de la représentation du personnel de La Poste.

du Cogas. Les autres dispositions de la proposition de loi concernant les droits syndicaux ou la protection des salariés détenant un mandat électif au sein d'une IRP correspondent peu ou prou à notre conception d'un rapport équilibré entre les employeurs et les employés. Néanmoins, nous devons rester vigilants pour que la centralisation associée à la mise en place des CSE ne soit pas synonyme d'une perte de proximité des représentants du personnel vis-à-vis des salariés et des enjeux directement associés au travail.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte, essentiellement technique, vise à appliquer à La Poste, premier employeur en France après l'État, la réforme du dialogue social que nous avons votée en 2017, favorisant et simplifiant l'exercice des responsabilités syndicales au moyen d'une nouvelle organisation. Des comités sociaux et économiques ont été créés pour fusionner les missions précédemment confiées aux délégués du personnel, aux CHSCT CHSCT et aux comités d'entreprise. Suivant ce modèle, une fusion des comités techniques et des CHSCT au sein des CSE a été opérée pour la fonction publique en 2019.

et son régime de représentation du personnel, défini en 1990, était celui d'une entreprise publique. Depuis lors, le développement d'autres activités, notamment bancaires, l'a conduite à devenir une société anonyme, à partir de 2010,

Cette situation, qui ne tient pas compte d'une évolution majeure du dialogue social, n'a pas d'équivalent. Il ne serait donc pas judicieux de la laisser perdurer. La proposition de loi prévoit une période de transition, qui permettra à la société de préparer la réforme en préservant la qualité de son dialogue social. Les mandats actuels arrivant à échéance le 31 janvier prochain, les instances actuelles ne disposent plus de base légale à partir de cette date. Le texte initial prévoyait la prolongation des mandats jusqu'aux élections et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2024.

Ces échanges l'ont conduite à reporter la date de fin de mandat des élus actuels au 31 octobre 2024, afin de laisser davantage de temps aux négociations en cours. Je pense que ce nouveau délai est satisfaisant et qu'il n'y a pas lieu de le repousser davantage. D'ailleurs, comme l'a rappelé la rapporteure, les syndicats ont signé à plus de 54 % l'accord de méthode, ce qui devrait apaiser les inquiétudes formulées sur certaines La proposition de loi rend ensuite applicables à La Poste les dispositions du code du travail concernant notamment le droit syndical, la négociation collective et les institutions représentatives du personnel.

Bien évidemment, la proposition de loi veille à prendre en considération la situation particulière des fonctionnaires, puisqu'elle crée un organisme les représentant, le conseil des questions statutaires, qui pourra être consulté sur les projets de lois et de règlements. Par ailleurs, les commissions administratives paritaires sont maintenues pour traiter des questions d'ordre individuel. En matière de représentativité, la réforme, calée sur les dispositions du code du travail, sera plus exigeante, puisqu'elle fixe un seuil de 10 % des suffrages exprimés lors des élections aux CSE.

validé ce dispositif en 2017. La mise en place des CSE dans une société d'une telle ampleur, présente sur tous nos territoires, n'ira pas sans difficulté. En commission, notre rapporteure a rappelé plusieurs points de vigilance, parmi lesquels l'enjeu de la proximité, tout particulièrement dans les territoires d'outre-mer.

Issue des relais de poste créés par Louis XI pour le transport des messages royaux, l'administration des postes en France trouve véritablement son origine au XVII siècle, avec la création de la poste aux lettres, dirigée par le surintendant général des postes.

l'emploi, à la fois, de fonctionnaires régis par des statuts particuliers, de salariés de droit privé et d'agents contractuels de droit public.

Or la loi du 6 août 2019 de transformations de la fonction publique disposait que les dispositions du code du travail relatives aux CHSCT continueraient à s'appliquer à La Poste jusqu'au prochain renouvellement des IRP. Néanmoins, aucune

L'article 2 de la proposition de loi instaure les comités sociaux économiques à La Poste ; là encore, je me réjouis que la commission ait reporté au 31 octobre 2024 la date butoir de leur mise en place. Enfin, son article 3 prévoit d'appliquer à La Poste, à titre transitoire, des dispositions du code du travail en vertu desquelles l'entreprise et les organisations syndicales pourront préparer la mise en place des CSE et l'organisation des élections professionnelles. Madame la ministre, mes chers collègues, l'instauration de comités sociaux et économiques à La Poste constitue un chantier à la fois vaste et complexe en raison de la diversité des statuts de son personnel. Le groupe Les Indépendants

ne doit pas ajouter à la complexité intrinsèque de ce projet. Prévoir une date d'application fixe constitue un élément de sécurisation du processus. Il convient par ailleurs que cette date corresponde à une année civile, pour des questions budgétaires liées notamment à la clôture des comptes du Cogas. Quel est l'avis de la commission

ce délai me semble suffisant pour mener les négociations sociales qui permettront de définir l'architecture des futurs CSE et les modalités d'organisation des élections professionnelles. Par ailleurs, il me semble important de préciser qu'un report jusqu'à la fin de décembre 2024 ne semble ni nécessaire ni souhaitable, alors que l'activité des mois de novembre et de décembre est très soutenue à La Poste. une prorogation trop longue des mandats des élus pourrait constituer une atteinte disproportionnée au droit d'expression des salariés. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable

Au fond, ce sont les protocoles d'accords électoraux qui vont définir les modalités d'organisation des élections aux CSE et qui peuvent ainsi déterminer leurs dates. Proroger les mandats jusqu'à la proclamation des résultats aux élections des CSE et au plus tard jusqu'au 31 octobre

Mme Corinne Féret. Cette proposition de loi impose un passage direct aux IRP de droit commun sans période transitoire « pédagogique ». Cela aboutit à faire subir un choc culturel et social aux personnels de La Poste. Plus de mille représentants syndicaux verront ainsi leur détachement prendre fin avec l'instauration des CSE. Cet amendement vise donc à prévoir un cadre pour la reconversion professionnelle de ces salariés, nécessaire à la mise en oeuvre d'une véritable gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Quel est l'avis de

outre, il appartient à La Poste de répondre à la question de la reconnaissance des compétences acquises par les représentants du personnel et de la valorisation de leur parcours, à savoir la possibilité d'évoluer du rôle de représentant vers un rôle de salarié ou de fonctionnaire classique.

certaines dispositions du code du travail trouveront à s'appliquer, notamment en matière de droit syndical et de protection des salariés concernés, afin de permettre aux organisations syndicales, ainsi qu'à l'employeur, d'organiser concrètement les élections des représentants du personnel aux CSE. Dans le même temps, les règles liées au statut particulier de La Poste continueront à

du dialogue social, sur la valorisation des parcours syndicaux. Elle permettra également l'adaptation et l'acclimatation des acteurs du dialogue social de La Poste à ce nouveau régime de droit commun, sans qu'il soit nécessaire de prévoir de nouvelles adaptations transitoires une fois ces CSE mis en place. L'avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement.

de loi prévoit en outre d'instituer un organisme représentant les fonctionnaires, qui sera consulté sur les questions statutaires. Rappelons que son organisation et son fonctionnement seront fixés par décret en Conseil d'État. Il ne me paraît donc pas nécessaire, ma chère collègue, de créer des instances supplémentaires. La commission a donc émis un avis défavorable

afin de prendre en compte la spécificité des territoires ultramarins, en garantissant que chaque collectivité ultramarine sera couverte par un CSE propre.

la mise en place d'un CSE est liée à la définition des établissements distincts au sein de l'entreprise, qui relève de la négociation collective ; elle n'est pas liée au découpage administratif des collectivités territoriales. Cela rend donc cet amendement difficilement opérationnel. Même si la proximité de la représentation est un enjeu de la réforme, tout spécialement dans les outre-mer, il revient aux partenaires sociaux de l'entreprise de définir le bon maillage de ces instances. Faisons confiance au dialogue social, faisons confiance aux syndicats qui ont soulevé cette problématique de la proximité,

notamment en prévoyant que la validité desdits accords est subordonnée à leur signature par toutes les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national.

à la mise en place des CSE et à l'organisation des élections professionnelles.

Les CHSCT étant dotés de la personnalité morale, il est nécessaire de prévoir le transfert de leurs droits et obligations aux CSE qui leur succéderont au sein de La Poste. Cet amendement vise donc à ce que l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des CHSCT

Le scrutin est clos. l'ensemble de la proposition de loi visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste.

la souffrance d'une planète à bout de souffle, nous courons à la catastrophe ». C'est ainsi qu'à la fin de son second mandat présidentiel Jacques Chirac nous parlait de la révolution écologique. Il nous reste toujours à l'accomplir

Tout d'abord, je remercie mes collègues coauteurs et cosignataires de cette proposition de loi. Nous avons eu des échanges fondamentaux durant sa construction. Ensuite, Ensuite, je remercie la commission des affaires économiques pour son important labeur sur le texte et tout particulièrement son rapporteur, Franck Menonville, qui a effectué un travail remarquable. En tant qu'agriculteur, il est imprégné des problématiques des territoires et connaît parfaitement celles du monde agricole, ce qui est un atout pour ce texte. Avant de vous parler de la proposition de loi, je reviendrai sur un point dont l'importance rythme, depuis le début de ma carrière, mon engagement politique : l'initiative parlementaire. Députés ou sénateurs, nous connaissons les besoins de nos territoires et de nos concitoyens. Nous avons la chance formidable d'être au contact des élus, des entreprises, des associations et de l'ensemble des entités faisant vivre nos territoires.

La France doit faire face à trois défis majeurs. Notre dépendance énergétique n'a jamais été aussi bien illustrée que dans la période actuelle. La guerre en Ukraine nous rappelle simplement ce que nous savions déjà : pour être souverains, nous devons être indépendants. Notre agriculture est en crise à de multiples niveaux. Notre souveraineté alimentaire est un gage de notre indépendance. Nos agriculteurs souffrent, mais l'agrivoltaïsme pourrait leur apporter un revenu complémentaire permettant de sauver leurs exploitations et d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. La France est également engagée dans une lutte contre l'artificialisation des sols. Ce n'est un secret pour personne : nous consommons des dizaines de milliers d'hectares par an. C'est vertigineux Ces trois problématiques sont intrinsèquement liées au dérèglement climatique. Nous devons faire évoluer notre bouquet énergétique en privilégiant le recours aux énergies bas-carbone. Notre agriculture va devoir s'adapter aux aléas climatiques. Nous devons réduire l'artificialisation des sols, car elle participe grandement à l'accélération du dérèglement L'agrivoltaïsme est une solution intéressante, qui n'artificialise pas les sols, mais participe à la production d'énergies renouvelables et apporte un revenu complémentaire à nos agriculteurs.

Je souhaite partager avec vous un exemple marquant : la Californie va installer des panneaux solaires sur des canaux d'irrigation afin de limiter l'évaporation de l'eau. L'objectif est impressionnant : sauver 286 milliards de litres d'eau chaque année ! La raréfaction de l'eau n'en finit pas de nous préoccuper. Le secteur agricole est l'un des plus grands consommateurs d'eau. Imaginons les effets positifs de l'agrivoltaïsme ! Il nous fallait une définition claire et un cadre précis.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est utile et nécessaire.

Le texte, après son passage en commission, est composé d'une dizaine de dispositions visant à encourager les projets alliant véritablement production agricole principale et production électrique secondaire, tout en prévenant le risque de conflits d'usages et l'essor incontrôlé de projets alibis. Pour ce faire, la proposition de loi, telle qu'adoptée à l'unanimité par notre commission, emporte plusieurs évolutions. crée d'abord un objectif de développement des installations agrivoltaïques, en réservant la priorité à la production alimentaire et en veillant à l'absence d'effets négatifs sur le foncier et sur les prix agricoles. Elle définit les installations agrivoltaïques comme des installations solaires permettant de maintenir ou de développer l'activité agricole. Ces installations doivent garantir une production agricole principale et un revenu durable en étant issu.

ensuite pour les installations agrivoltaïques une obligation d'achat et une procédure de mise en concurrence spécifique. Elle permet aux parcelles agricoles présentant de telles installations de bénéficier des aides de la politique agricole commune Enfin, elle clarifie la procédure d'autorisation d'urbanisme prévue pour les installations agrivoltaïques, en prévoyant un avis systématique de la Un autre garde-fou est la constitution de garanties financières pour assurer le démantèlement et la remise en état des sites, préservant ainsi la réversibilité des Notre commission a veillé à enrichir le texte, en adoptant une dizaine d'amendements visant à préserver les intérêts agricoles et les compétences locales. Ainsi, la définition de l'agrivoltaïsme a été clarifiée pour tenir compte des travaux consensuels de l'Agence

Ces enrichissements, qui nous permettent aujourd'hui de disposer d'un texte équilibré et cohérent, n'ont été possibles que grâce au travail effectué en bonne intelligence avec notre collègue Jean-Pierre Decool, auteur de la proposition de loi, que je félicite vivement.

Cette filière peut être porteuse d'externalités positives pour nos agriculteurs, en leur offrant un complément de revenu et une protection contre certains aléas, notamment climatiques.

d'autant que les installations agrivoltaïques ne sont pas décomptées dans l'artificialisation des sols, de par une disposition introduite par notre commission dans la loi du 22 août 2021 à encadrer l'agrivoltaïsme, pour garantir que l'activité agricole demeure l'activité principale de la parcelle et ainsi prévenir les dérives que nous commençons parfois à observer dans nos territoires. Il entend aussi simplifier et encourager le développement de projets porteurs d'une réelle plus-value, qui sont nombreux. Enfin, il vise assurément à répondre au double objectif de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté énergétique. Le texte élaboré par notre commission s'inscrit ainsi dans la droite ligne des travaux antérieurs de simplification des normes en matière d'énergies renouvelables. Depuis 2020, pas moins de 30 solutions de simplification ont été adoptées par notre commission : 10 portaient sur l'hydroélectricité, 3 sur l'hydrogène,

Alors que le Président de la République a annoncé son souhait de promouvoir l'agrivoltaïsme, dans son discours prononcé à Saint-Nazaire le 22 septembre dernier, le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, délibéré en conseil des ministres le 26 septembre, est muet sur ce point. Je souhaite que le Sénat comble cet angle mort. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter largement cette proposition de loi. C'est une occasion unique de légiférer en amont sur un domaine d'avenir, en répondant à la fois aux besoins de soutien et de régulation.

il nous faut aujourd'hui trouver des solutions pour concilier souveraineté alimentaire et indépendance énergétique. Tel est, au fond, tout l'enjeu du débat que nous allons avoir sur cette proposition de loi inscrite à l'ordre du jour du Sénat sur l'initiative du groupe Les Indépendants - République et Territoires, que je remercie. La guerre en Ukraine, La guerre en Ukraine, qui affecte à la fois les marchés agricoles et énergétiques, illustre l'importance de traiter ces deux enjeux conjointement. La transition énergétique doit permettre de limiter la trajectoire de réchauffement climatique et de gagner autant en indépendance énergétique qu'en résilience, à la fois pour nos concitoyens et nos agriculteurs. nos agriculteurs. Ceux-ci sont les premiers à subir les effets croissants du dérèglement climatique dans nos territoires, mais ils sont également des acteurs à part entière de l'adaptation à ce changement. du climat (Giec) nous dit que nous pouvons encore inverser la tendance. Il faut pour cela reprendre en main notre destin énergétique, ce qui implique de remplacer 65 % de notre consommation d'énergie finale, qui vient encore aujourd'hui du bout du monde

Aucune des transitions à l'oeuvre- transitions nécessaires ! -ne pourra se faire sans notre agriculture. Nous ne le disons pas suffisamment : nos agriculteurs détiennent une partie de la réponse au problème de la lutte contre le réchauffement climatique. Ils portent au quotidien, dans tous nos territoires, des projets qui contribuent par la production d'énergies renouvelables qui se substituent aux énergies fossiles, comme les biocarburants ou la méthanisation. Les technologies agrivoltaïques permettent dans le même temps d'apporter des services aux agriculteurs, en protégeant davantage les cultures contre les aléas météorologiques, en régulant leur exposition au soleil, ou encore en les protégeant contre un excès de précipitations ou des épisodes de grêle.

De plus, en 2022, le Gouvernement a décidé d'étendre ce soutien en permettant aux porteurs de projets agrivoltaïques de répondre aux appels d'offres photovoltaïques sur les bâtiments. Cela a d'ores et déjà permis à de premiers projets d'émerger, dans les territoires, en concertation avec l'ensemble des acteurs impliqués. Cependant- et c'est la raison pour laquelle je considère que cette proposition de loi est très importante -, il est nécessaire d'aller plus loin pour accélérer et garantir le développement cohérent et maîtrisé de ces projets agrivoltaïques dans nos territoires.

avec les acteurs locaux- les maires au premier chef, mais aussi les agriculteurs, ou encore les chambres d'agriculture. C'est peut-être une évidence, mais l'agrivoltaïsme que nous promouvons va de pair avec la préservation de terres agricoles productives, essentielles pour notre souveraineté alimentaire. Je sais que le Sénat est particulièrement attentif à ces enjeux.

non-artificialisation des sols, conservation des fonctions écologiques et du pouvoir agronomique du sol, maintien d'une activité agricole significative, réversibilité totale des projets, capacité du préfet de contraindre à la constitution de garanties financières, avis systématique de la CDPENAF et, évidemment, service ajouté réel apporté à l'agriculteur. Ce cadre, ainsi posé, constitue un véritable progrès par rapport à la situation actuelle. Le Gouvernement considère que la définition proposée dans ce texte va véritablement dans la bonne direction, notamment grâce à un encadrement clair des projets permettant d'éviter tous les détournements. Un agriculteur doit rester un agriculteur et l'agrivoltaïsme doit rester de l'agrivoltaïsme ! Ces règles strictes permettront de lutter contre les projets alibis et contre les abus, tout en améliorant la sécurité juridique pour toutes les parties prenantes, et ainsi, d'accompagner le développement concerté de l'agrivoltaïsme.

notamment pour apprécier la synergie entre les deux activités- agricole et énergétique -, prendre en compte les spécificités des territoires et inscrire les projets dans la durée. Nous travaillons aujourd'hui pour les générations de demain ; cela nous oblige tous. Nous devons donc aussi penser à la transmission. En aval, les conditions de retour à l'activité agricole des surfaces sur lesquelles des installations agrivoltaïques auront été implantées doivent être anticipées. C'est l'enjeu de la réversibilité, qui est traitée dans cette proposition Se posent des questions de pérennité des investissements, notamment au moment de la transmission des exploitations, de solvabilité des installateurs à terme et de responsabilité. concernant l'éligibilité aux aides de la politique agricole commune, l'engagement du Gouvernement est clair : à partir du moment où l'agrivoltaïsme aura été défini avec précision et justesse dans la loi, nous définirons l'éligibilité des projets aux aides de la PAC. Cela suppose, toutefois, pour être en conformité avec le droit européen, d'avoir la définition la plus précise possible de l'agrivoltaïsme. C'est pourquoi il est important de s'en tenir précisément à la définition issue des issue des travaux de l'Ademe. Le plan stratégique national (PSN) de la France, approuvé le 31 août dernier par la Commission européenne, précise à cet égard que « l'admissibilité des surfaces couvertes par des panneaux photovoltaïques sera précisée dans la réglementation nationale ».

Voilà tracées les grandes lignes de ce débat. Je forme le voeu qu'il permette, en lien étroit avec les organisations professionnelles agricoles et avec l'ensemble des acteurs du monde rural- je pense en particulier aux élus -de préparer un dispositif équilibré en vue des débats à venir sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, 34 degrés à Orthez et 31 degrés à Biarritz ce mardi, 26 degrés à Nantes hier : un bon tiers sud-ouest de la France connaît actuellement des températures dignes d'un plein été.

Le réchauffement s'accélère. Cela donne raison au Giec, qui nous alerte sur l'augmentation exponentielle des températures et nous suggère des alternatives pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi limiter les conséquences du changement climatique.

Le Gouvernement est donc au travail, mais le Sénat n'est pas en reste, comme en témoigne cette proposition de loi. Le photovoltaïque fait en effet partie de la réponse.

Aujourd'hui, elle atteint quelque 10 gigawatts. Il faudrait donc installer, pour atteindre cet objectif, 3 à 4 gigawatts de panneaux solaires par an, contre 1 gigawatt aujourd'hui. Nous devons accélérer et trouver des possibilités d'installer du photovoltaïque. L'agrivoltaïsme fait partie des solutions qu'il faut saisir et encourager. La combinaison du solaire et des activités agricoles représente en outre un complément potentiel de revenus très important pour nos agriculteurs. Cela étant dit, cet encouragement ne doit pas être synonyme d'aveuglement. L'essor de l'agrivoltaïsme est réel dans nos territoires,

À cette fin, il impose un certain nombre de garde-fous : la réversibilité des panneaux, la destination principalement agricole de l'activité menée sur la parcelle, ou encore le caractère systématique de l'avis de la CDPENAF. Ce cadre vise à éviter toute spéculation énergétique. En d'autres termes, cette proposition de loi entend réguler une activité nécessaire à la décarbonation de notre énergie,

dans la production d'énergies renouvelables. En janvier dernier, lors de l'examen de la proposition de résolution sur le même sujet, nous avions déjà dénoncé un manque d'encadrement des risques liés à la croissance de cette activité. Notre raisonnement et nos constats sont les mêmes aujourd'hui, car la proposition de loi que nous examinons

L'émergence d'installations suscite déjà bien des inquiétudes, voire des oppositions, tant notre foncier agricole est déjà soumis à une pression croissante. L'installation de panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles emporte des risques multiples. Elle peut déséquilibrer les dynamiques économiques agricoles locales, artificialiser davantage les sols, compromettre l'installation de jeunes agriculteurs en accaparant le foncier, sans garantie de réversibilité ni de transmission des parcelles, porter atteinte à la biodiversité et à l'esthétique des paysages ; enfin, elle pourrait fragiliser notre souveraineté alimentaire par un glissement sournois, à terme, de ces surfaces vers la seule production d'énergie. La question du cadre réglementaire est donc fondamentale. À notre sens, elle s'articule selon cinq points, sur lesquels nous avons tenté d'apporter des réponses par voie d'amendement. Le premier concerne la définition des installations agrivoltaïques Pour être considérées comme telles et bénéficier pleinement à une exploitation agricole, tout en contribuant à nos objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050, ces installations doivent apporter au moins un service à l'exploitation : amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas, ou amélioration du bien-être animal. Une autre condition est qu'elles soient réversibles. La priorité doit être accordée à la production alimentaire ; aussi les parcelles converties en agrivoltaïsme doivent-elles pouvoir retourner à leur vocation d'origine si nécessaire. d'un point de vigilance majeur ; nous avons donc déposé un amendement visant à rendre automatique la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état d'un site pour les projets dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 Le deuxième point porte sur le contrôle des installations et de leur financement. Cette question incontournable est sans doute l'une des plus difficiles à résoudre, dans la mesure où elle touche aux finances publiques. Une fois les installations autorisées et mises en service, qui veillera au respect des critères que je viens d'énoncer, notamment à l'apport des services ? Avec quels moyens humains et financiers ? Dans un souci de préservation de l'activité agricole, il faut introduire des dispositions de suivi et de contrôle, ainsi que des possibilités de démantèlement en cas de non-respect de la loi. L'absence de contrôles opérés par l'État donnera lieu sans aucun doute à des dérives ; nous nous y opposons.

Nous avons formulé cette proposition par voie d'amendement, afin que les communes soient toujours informées en amont lorsqu'un groupement propose la réalisation d'un projet agrivoltaïque sur leur territoire. À cet égard, nous tenons à souligner que la répartition de la fraction de l'imposition

Il est également impératif de réfléchir aux modalités de transmission, dans le cas d'un exploitant fermier comme dans celui d'un exploitant propriétaire. Le repreneur, en pleine propriété ou en fermage, doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages que l'exploitant actif au moment de la mise en place des installations agrivoltaïques. Nous formulons donc les propositions suivantes : il convient de subordonner la qualification d'agrivoltaïsme à celle d'agriculteur actif et d'encadrer la transmission des parcelles en agrivoltaïsme, notamment en prévoyant les conditions du départ à la retraite ou de la cessation d'activité de l'exploitant dans le contrat initial. Il s'agit selon nous de garanties indispensables pour éviter une artificialisation masquée et assurer une transmission réussie de ces parcelles. Notre principale ligne directrice est d'éviter à tout prix que notre autonomie alimentaire et notre autonomie énergétique n'entrent en conflit

En janvier dernier, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s'était abstenu lors de l'examen de la proposition de résolution sur le même thème en séance publique, estimant que le sujet du développement de l'agrivoltaïsme nécessitait de mettre en place « des garde-fous afin de prévenir toute dérive irréversible sur notre modèle agricole » et de ne pas favoriser l'émergence « d'énergieculteurs Nous avions néanmoins souligné que nous étions disposés à accompagner le développement de l'agrivoltaïsme, dès lors qu'il s'agirait bien de techniques ayant d'abord pour but d'améliorer la production agricole et non de l'utiliser comme alibi au profit d'une production plus rentable.

car il n'existe pas aujourd'hui de définition précise de l'agrivoltaïsme. Ce manque s'accompagne de dérives et de conflits d'usages auxquels il faut impérativement apporter une réponse. En effet, alors que 18 % des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté et qu'un tiers seulement de leurs revenus est issu de l'agriculture, l'énergie solaire prend des airs de nouvel or vert pour des agriculteurs qui ont de plus en plus de mal à vivre de leur activité. C'est pourquoi il est impératif de réaffirmer la vocation nourricière des terres agricoles et la priorité de la production alimentaire sur la production énergétique. Cela est vrai pour le développement de toute forme d'énergie : photovoltaïque, méthanisation, etc. Comme le rappelait mon collègue Gérard Lahellec, qui a été membre de la mission d'information sur la méthanisation dans le mix énergétique, nous assistons aujourd'hui à une guerre entre éleveurs laitiers et méthaniseurs. Les premiers peinent à nourrir leurs troupeaux et à obtenir un prix rémunérateur pour leurs productions et leur lait ; les seconds sont incités à accélérer leurs investissements pour produire davantage de gaz vert. Avec la crise énergétique que nous traversons, le débat s'exacerbe autour des objectifs de production de biogaz et nous devons sans cesse poser ces questions fondamentales : quelle agriculture voulons-nous ? Quels écueils devons-nous éviter afin d'empêcher que notre agriculture ne vise que des objectifs purement industriels, souvent plus rémunérateurs que sa finalité première, qui est et doit rester l'alimentation ? En ce sens, la question du revenu paysan ne se résoudra pas par la multiplication des revenus complémentaires, voire des revenus Pour autant, nous saluons le travail des auteurs de la proposition de la loi et du rapporteur. En effet, l'agrivoltaïsme peut être un outil agricole ayant pour but premier de protéger les cultures de températures extérieures trop fraîches ou trop élevées ainsi que de la grêle, voire de réduire la consommation d'eau.

ou de développer l'activité agricole, « en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en veillant à l'absence d'effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ». De même, la notion de réversibilité, proposée par l'Ademe, a été introduite dans le texte en commission.

je tiens tout d'abord à saluer l'auteur de cette proposition de loi et le travail effectué par le rapporteur. Les amendements de ce dernier ont largement contribué à rapprocher ce texte de la proposition de résolution

La diminution des terres arables est continue dans notre pays depuis le milieu des années 1950 et notre agriculture connaît des difficultés nouvelles auxquelles il nous faut apporter La souveraineté alimentaire ne doit donc pas être troquée contre la souveraineté énergétique. Malgré quelques différences de forme sur ce texte, qui ont donné lieu au dépôt d'amendements par notre groupe, nous sommes très majoritairement satisfaits de l'équilibre trouvé.

prévoit l'apport de services agronomiques ou écologiques sur les surfaces où l'agrivoltaïsme est implanté. Ce prérequis nous semble tout à fait justifié, dans la mesure où l'agrivoltaïsme ne peut se résumer à un photovoltaïque classique, qui viendrait se superposer aux cultures sans prendre en compte leurs spécificités. Nous maintenons, malgré notre soutien à cette proposition de loi, que les installations photovoltaïques doivent être placées en priorité sur des surfaces déjà urbanisées et artificialisées. Cet argument est d'autant plus valable que, dans quelques jours, notre assemblée examinera un projet de loi portant sur l'accélération de la production d'énergies renouvelables, qui prévoit l'équipement obligatoire des parkings. L'équipement massif de zones déjà artificialisées doit nous conduire à une sélectivité accrue des projets d'équipements sur des zones non artificialisées, comme les surfaces agricoles.

Le soutien public financier apporté aux projets la procédure de guichet ouvert, tel qu'il est inscrit dans ce texte, nous semble disproportionné. Il pourrait conduire, dans certaines conditions définies par cette proposition de loi, à soutenir des projets de taille importante, allant jusqu'à six mégawatts, voire au-delà, lesquels pourraient pourtant être rentables dans des conditions de marché. Il nous semble inopportun de soutenir dans une trop large mesure de tels projets, qui doivent trouver un équilibre économique par eux-mêmes et n'ont pas besoin d'argent public pour voir le jour. Enfin, plusieurs amendements de notre groupe visent à perfectionner ce texte, en particulier sur le sujet du mécanisme de compensation agricole, auquel les projets agrivoltaïques pourraient légitimement être soumis, au même titre que les projets photovoltaïques classiques. Nous formulons également des propositions concernant les provisions pour frais de démantèlement des installations et le suivi statistique des implantations agrivoltaïques.

N'aurait-il pas été plus logique d'analyser les enjeux, d'établir un diagnostic des risques et de réunir autour d'une table l'ensemble des parties prenantes avant de lancer les projets ? Il faut dire que les entreprises ont toujours une longueur d'avance en matière de stratégie et qu'elles savent flairer les opportunités économiques ! Quels sont les enjeux ?

de répondre au projet ambitieux d'atteindre 40 % d'énergie renouvelable d'ici à 2030 en France. C'est précisément cet objectif qui a suscité l'engouement des sociétés d'énergie pour notre foncier agricole, une opportunité qui leur coûte peu, mais qui présente un risque

L'installation photovoltaïque doit ainsi apporter un service en réponse à une problématique agricole. » Je suis allé visiter une installation photovoltaïque sur une exploitation viticole dans le Vaucluse et j'ai bien compris le service rendu en matière de protection contre la grêle, grâce à des filets intégrés aux panneaux,

des porteurs, peu de paysans pouvant assumer eux-mêmes le coût de ces installations très onéreuses. C'est pourquoi je défendrai un amendement qui vise à écarter de l'agrivoltaïsme toute installation qui ne permettrait pas de garantir « un partage équitable de la valeur générée par la production énergétique entre l'exploitant agricole et les autres acteurs du projet

Comment empêcher des agriculteurs de choisir cette voie alors que d'autres s'y sont déjà engouffrés ? Cela ne serait pas juste. Les amendements que nous allons défendre ont pour objectif de sécuriser les agriculteurs en insistant sur la notion d'activité agricole majoritaire, la production d'électricité ne doit être qu'une activité secondaire. L'agrivoltaïsme ne doit pas non plus faire de l'ombre au photovoltaïque sur les toits et sur les friches.

remercions Jean-Pierre Decool pour sa proposition de loi, qui rappelle d'abord toute la responsabilité des parlementaires. Sa conviction est unanimement partagée dans cet hémicycle

lors que l'on sort de l'anecdotique et que le sujet concerne des milliers de communes françaises, ce débat va nous éclairer sur les conditions d'autorisation au regard du droit de l'urbanisme.

un avis, rarement compréhensif et positif, sur la perspective d'avoir comme voisinage un, deux, voire trois hectares de panneaux photovoltaïques. Il faudra donc expliquer et

Le groupe Les Républicains va voter ce texte, parce qu'il permet d'avancer. Il ne réglera pas tout : l'enjeu touche à la coexistence de l'électrique et de l'agricole,

toutefois une idée : le monde rural participe au développement des activités d'énergies renouvelables. Or, entre la location du sol-

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis quelques mois, la crise ukrainienne nous rappelle l'urgence de plus en plus brûlante de notre indépendance énergétique.

Les installations photovoltaïques s'inscrivent dans cette évolution. Parmi elles, l'agrivoltaïsme apparaît comme un domaine prometteur qu'il serait regrettable de ne pas exploiter, et ce pour plusieurs raisons.

La lutte contre l'artificialisation des sols oblige à employer des procédés innovants. Ensuite, de nombreuses études montrent le bénéfice direct de l'agrivoltaïsme pour la biodiversité et les cultures, grâce aux effets des ombrières et à la limitation de l'évaporation d'eau, qui améliorent nettement certains rendements. Enfin, et à condition de veiller au maintien des aides de la PAC et aux garanties de rachat de l'électricité sur ces parcelles, ce dispositif est capable de générer des revenus complémentaires pour les agriculteurs, qui en ont grand besoin. Les disparités climatiques et topographiques de notre pays sont nombreuses et sources de situations économiques et agricoles très diverses en fonction des secteurs. Il en va de même des disparités des aides liées à la PAC en fonction des zonages. Pour autant, quelle que soit la zone concernée, le développement de l'agrivoltaïsme fait naître de réels espoirs et des attentes, particulièrement dans les territoires situés au sud de la Loire, régions trop souvent oubliées au moment de la distribution de certaines enveloppes. Lors de nos travaux précédents, nous avions pointé des problématiques essentielles au développement de l'agrivoltaïsme, notamment celles du maintien de la PAC, des autorisations administratives, des contrats de rachat, ou encore de la fiscalité appliquée. Ce texte a vocation à y répondre.

qui prévoit des mesures transitoires de facilitation et de simplification des procédures d'études des projets nécessaires à notre transition énergétique. On nous propose pour une fois de desserrer l'étau des contraintes légales et réglementaires. N'ayons pas peur de cette liberté Évitons les complexifications à outrance et l'inflation d'amendements qui, en visant une exhaustivité impossible, auraient pour conséquence de nous éloigner du coeur du problème et donc de sa solution. Il ne s'agit ni de légiférer à la va-vite ni d'inonder les territoires de panneaux photovoltaïques, mais de rester vigilants et pragmatiques quant à l'encadrement de la définition de l'agrivoltaïsme

Je tiens à remercier tous ceux qui ont enrichi ces travaux de leur participation et de leur réflexion, en particulier les coauteurs de la proposition de loi, le groupe Les Indépendants - République et Territoires, notre excellent rapporteur et les services de la commission des affaires économiques. Souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire, tel est le double bénéfice que nous voyons dans cette proposition de loi, dont notre groupe est fier de se faire le porte-voix.

condition toutefois qu'il réponde à un certain nombre de critères auxquels il ne pourra déroger. À l'heure où les projets se développent à grande vitesse dans les territoires, il devient urgent de mettre en place un cadre précis et une stratégie lisible pour les acteurs concernés on accompagnera le déploiement régulé d'un agrivoltaïsme vertueux. C'est pourquoi nous saluons l'objectif des auteurs de cette proposition de loi : fixer un cadre juridique et budgétaire à l'agrivoltaïsme.

ni laisser s'installer une concurrence potentiellement déloyale entre production alimentaire et production non alimentaire. L'agrivoltaïsme doit être un facteur d'amélioration de la production agricole principale, en synergie avec une production énergétique qui doit rester secondaire. En parallèle, le maintien ou l'amélioration des revenus agricoles doit être assuré. De plus, il nous faut veiller à ce que ces installations respectent scrupuleusement les normes en matière d'urbanisme, de patrimoine et de paysages. L'avis conforme de la CDPENAF nous semble là aussi indispensable et apparaît comme un outil stratégique pour ajuster les projets en fonction des réalités des territoires et des besoins des agriculteurs. le risque d'artificialisation des terres. Les ancrages en béton, les clôtures, les lignes électriques enterrées et les voies d'accès peuvent affecter les sols ou perturber la faune et la flore. Il faut investir dans des installations matériellement réversibles ; nous saluons l'ajout effectué sur ce point,

Cette définition doit fournir toutes les garanties nécessaires à la protection de la biodiversité et au maintien de la vocation nourricière des terres et des services écosystémiques des sols. Il convient, en ce sens, de distinguer le photovoltaïque au sol et l'agrivoltaïsme. Quand le premier a pour unique vocation la production d'énergie et peut contribuer à l'artificialisation des sols, le second devrait, selon la définition qui serait actée dans le code de l'énergie, apporter un service à une problématique agricole et contribuer à une certaine résilience vis-à-vis du changement climatique, à l'heure où les agriculteurs sont les premiers touchés. Si la définition proposée par le rapporteur nous paraît aller globalement dans le bon sens, nous défendrons toutefois un amendement visant à renforcer encore davantage les garde-fous, notamment sur le revenu agricole et sur la transmission des parcelles. La succession, comme je l'ai indiqué précédemment, nous semble en effet un enjeu fondamental. Ce texte a le mérite de poser un cadre juridique et une orientation stratégique. Notre vote dépendra toutefois de l'adoption ou non d'un certain nombre de dispositions qui nous paraissent primordiales. La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

L'agrivoltaïsme suscite autant d'engouement que de divisions, à raison. Le sujet se situe en effet au coeur de deux enjeux majeurs, celui de la souveraineté alimentaire et celui de la souveraineté énergétique.

L'agrivoltaïsme répond à deux objectifs : apporter un complément de revenu à nos agriculteurs et permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs en matière de développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque d'ici à 2028. Ces objectifs sont compris entre 35,1 et 44 gigawatts. Toutefois, à la fin du troisième trimestre 2021, notre pays ne compte que 12,3 gigawatts d'installations photovoltaïques et l'on estime qu'il 33 000 et 44 000 hectares d'installations de ce type pour atteindre les objectifs de notre programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous sommes donc en retard et les terres agricoles offrent bien une option supplémentaire qu'il nous faut considérer,

Atteindre nos objectifs énergétiques doit être une priorité au moment où notre pays fait face à une crise énergétique majeure, mais il ne faut pas le faire de manière anarchique. pas plus tard que la semaine dernière, le journal révélait que le gouvernement britannique s'interrogeait sur la nécessité de durcir les modalités d'installation des panneaux solaires sur les terres agricoles.

et l'obligation de fournir au moins un service à l'environnement. En vertu de cette définition, la notion d'activité agricole principale devra pouvoir être appréciée au regard de l'emprise au sol, de la production ou du revenu. La commission a également renforcé le pouvoir des élus en supprimant l'autorisation de principe d'installation des projets agrivoltaïques et en renforçant la territorialisation des projets, notamment l'information préalable des élus locaux pour tout projet d'installation agrivoltaïque. Ces modifications vont dans le bon sens. L'examen de cette proposition de loi s'inscrit dans un calendrier très particulier, puisque nous examinerons dès la semaine prochaine en commission et le 2 novembre en séance publique le très attendu projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

nous donne donc l'opportunité de mener un travail de réflexion préalable et de poser les bases d'une définition de l'agrivoltaïsme et d'un encadrement juridique pérenne. Aussi, je souhaite que nous puissions profiter de ces échanges pour trouver un consensus et un équilibre acceptable afin de permettre un développement contrôlé

Pour ma part, je considère que légiférer sur l'agrivoltaïsme, c'est mettre un pied dans la porte pour crédibiliser la compétition entre l'agriculture nourricière et la production énergétique. Notre rôle de législateur est de préserver la vocation nourricière de la terre et ainsi la raison d'être des agriculteurs. Vous pouvez tous constater, mes chers collègues,

Ne nous y trompons pas, les installations d'agrivoltaïsme se feront à proximité des villes et des métropoles, là où les besoins énergétiques sont les plus importants, mais aussi là où l'autonomie alimentaire est la plus faible- avec un niveau proche de 2 % -, et non pas obligatoirement là où un complément de revenu pour les par l'Ademe en 2018, le potentiel d'installation de panneaux photovoltaïques sur les grandes toitures, sur les friches industrielles et sur les parkings permet largement d'atteindre l'objectif de 100 gigawatts pour l'énergie photovoltaïque qu'a fixé le président de la République.

nous avons de nombreuses interrogations, voire des inquiétudes, comme j'ai pu le rappeler dans la discussion générale. En tout état de cause, en déposant une dizaine d'amendements, notre groupe ne souhaite nullement faire obstruction ; nous avons bien conscience que nos collègues du groupe Les

et quand on est vieux, on souhaite qu'il soit élevé, pour pouvoir financer sa cessation d'activité. Par conséquent, je ne comprends pas la rédaction de cet amendement. C'est la raison pour laquelle je me rallierai à la position

et rend la cession ou l'acte de vente beaucoup plus compliqués, en particulier pour les agriculteurs dont les revenus sont limités, qui connaissent souvent des difficultés

Le texte issu des travaux de la commission prévoit « un maintien et un développement » de la production agricole dans le cadre de l'installation de systèmes agrivoltaïques, mais les critères permettant de définir ce maintien apparaissent insuffisamment exigeants au regard de l'enjeu de protection de la vocation agricole des surfaces concernées. Mon amendement vise donc à consacrer plusieurs

texte de la commission. En second lieu, en proposant une rédaction globale, l'amendement écraserait les garde-fous introduits par la commission pour encadrer l'agrivoltaïsme. Je demande donc son retrait,

Nos amendements l'illustrent : la définition législative de l'agrivoltaïsme et, partant, la distinction entre les pratiques à encourager et celles à freiner ne font pas l'objet d'un consensus ; à ce jour, cette définition manque de clarté. Le texte que nous examinons propose d'abord une description de l'installation agrivoltaïque, puis une définition positive et une définition négative, le tout devant être précisé par décret. Cette complexité présente autant de risques juridiques. Le texte de la commission prévoit notamment que l'installation devra apporter directement à la parcelle au moins un service, tout en garantissant « une production agricole significative et un revenu durable en étant issu.

Quant aux revenus énergétiques, ils pourraient dissuader les agriculteurs d'exercer leur métier originel, ce qui ne permet pas de mettre un frein au développement des projets alibis. C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement, qui vise à remplacer les notions de « production agricole significative » et de « revenus durables en étant issu », qui posent des difficultés pour la majorité des acteurs auditionnés, par des critères liés à l'absence de dégradation importante de la qualité et de la quantité de production agricole, ou de diminution des revenus issus de cette production, à l'instar de la définition proposée par l'Ademe. L'adoption de cet amendement permettrait de prendre en considération la qualité de la production agricole et de préserver la vocation actuelle des terres.

Cet objectif peut rejoindre celui « d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques », déjà présent dans la liste des services pouvant être apportés par l'installation. Nous pouvons comprendre la nécessité de renvoyer à un décret la définition précise de ces services à atteindre

de l'Ademe. Or la protection des cultures agricoles contre les aléas climatiques constitue l'un des grands apports de l'agrivoltaïsme. En effet, dans le cadre de l'agrivoltaïsme dit « dynamique », des start-up, notamment sur mon territoire, apportent des solutions révolutionnaires, grâce à des panneaux solaires modulables et pilotables par l'agriculteur

dont il convient de protéger les parcelles agricoles. Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à évoquer expressément les aléas météorologiques. Les deux

être fournis à la parcelle agricole, en y incluant des services dits « indirects », afin d'adapter les types de projets à la réalité des exploitations. Les développeurs doivent pouvoir atteindre ces objectifs en concertation avec les agriculteurs. Les critères additionnels proposés dans cet amendement sont la contribution à la transition agricole, le maintien ou l'amélioration de la biodiversité, ainsi que l'amélioration de l'écosystème agricole et l'utilisation durable des sols. L'amendement

des services devant être rendus par une installation agrivoltaïque pour qu'elle soit considérée comme telle. À l'heure du changement climatique et de la chute dramatique de notre biodiversité, comme le précisent les derniers rapports de la insérer un objectif de maintien ou d'amélioration de la biodiversité est indispensable. Il semblerait fortement regrettable, si ce n'est inconcevable, qu'une installation agrivoltaïque vienne dégrader la biodiversité environnante. Or les quatre services retenus dans le présent article n'assurent pas une prise en compte spécifique de cet

La commission a souhaité qu'un décret, pris après consultation des acteurs agricoles, vienne définir ces termes. Elle a précisé que la production agricole principale Elle a précisé que la production agricole principale pourra ainsi être déterminée au regard- c'est un ajout de la commission des affaires économiques -du volume de production, du niveau de revenu et de l'emprise au sol.

L'amendement n° 4, comme son objet l'indique, est déjà satisfait par le premier critère de service rendu par une installation agrivoltaïque. Par ailleurs, la définition de l'Ademe, que la commission a souhaité retenir et renforcer,

donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Une exploitation agricole est une aventure personnelle, une aventure économique ; c'est l'histoire d'une vie, le résultat de choix responsables faits par des femmes et des hommes

Devésa. Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit qu'une installation agrivoltaïque ne peut pas porter une atteinte substantielle ou limitée aux services listés : amélioration du potentiel et de l'impact agronomique ; adaptation au changement climatique ; protection contre les aléas

Le législateur doit se montrer aussi ambitieux que les forces vives de notre pays, prêtes à pousser plus loin le curseur en faveur d'une agriculture nouvelle. Il conviendrait ainsi de considérer qu'une installation agrivoltaïque ne peut porter atteinte à aucun des critères de définition mentionnés ci-dessus, ni substantiellement ni limitativement. L'amendement

ou une atteinte limitée à deux d'entre eux. Le présent amendement vise à renforcer ce dispositif, en prévoyant qu'une installation ne pourra pas porter atteinte de façon substantielle à au moins deux services et de façon

l'amendement n° 39 conduirait à retirer les précisions utiles, initialement apportées par l'auteur de la proposition de loi, concernant les atteintes aux services pouvant être rendus par une installation agrivoltaïque. L'équilibre trouvé par l'auteur de ce texte, voulant qu'une installation portant une atteinte substantielle ou deux atteintes limitées à un service ne puisse pas être qualifiée d'agrivoltaïque, est un bon compromis. Il permet, d'une part, de sécuriser la définition, les projets

les notions de « substantielle » et de « limitée », qui seront utilement précisées par décret, pour ne conserver que la notion d'« atteinte » de manière générale, risque de conduire à des débats sans fin sur le niveau d'atteinte acceptable engendrée par une installation agrivoltaïque.

Les installations agrivoltaïques pourraient engendrer des revenus significatifs, dont une partie devrait pouvoir ruisseler jusqu'à l'agriculteur qui leur consacre des terres de son exploitation. Les revenus doivent donc être équitablement partagés.

je le retire,

Il s'agit de veiller à ce que cette activité ne devienne pas le prétexte à une production d'énergie, même si cette dernière est renouvelable, vertueuse, et s'inscrit dans les objectifs nationaux et européens de développement des énergies renouvelables. C'est pourquoi, dans le cadre du futur décret mettant en oeuvre ce texte, la production agricole et les revenus qui en sont issus doivent rester prépondérants.

prépondérant de la production et du revenu agricoles, proposée dans cet amendement, n'est pas opportune pour deux raisons. Tout d'abord, elle est redondante avec le reste de la définition. Ensuite, une telle précision exclurait de la définition des agriculteurs pouvant rencontrer des difficultés de production ou de revenu, mais aussi certaines surfaces destinées à des productions à faible valeur ajoutée.

principale doit- et non peut -s'apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu et de l'emprise au sol. Dans la continuité des amendements précédents, les sénateurs socialistes souhaitent lutter contre les effets d'aubaine et mettre en place des garde-fous pour éviter que l'activité agricole ne devienne une excuse à la production d'énergie.

D'une part, elles supprimeraient le pouvoir d'appréciation tant des services déconcentrés de l'État que des acteurs agricoles, dans la définition réglementaire de la notion d'activité agricole principale. Or les acteurs de terrain eux-mêmes sont les mieux placés pour convenir de la définition la plus adaptée. la modification suggérée réduirait à trois le nombre de critères pouvant être inclus dans cette définition, alors que d'autres critères pourraient être utiles le cas échéant : le statut de l'agriculteur, le partage de la valeur, ou encore l'enjeu de la transmission. Nous perdrions donc

du 2 décembre 2021 sur la politique agricole commune peut servir de point de référence pour déterminer réglementairement la notion d'activité agricole principale.

? Vous souhaitez lier les notions d'agrivoltaïsme et d'activité agricole principale à la réglementation relative aux aides de la PAC. D'abord, rappelons que toutes les parcelles agricoles ne sont pas soumises aux règles d'admissibilité des aides de la PAC. Je pense en particulier à la filière viticole, où de nombreux viticulteurs ne demandent pas ces aides. Compte tenu des règles spécifiques prévues dans la réglementation européenne et déclinées dans le plan stratégique national, il n'est pas opportun de traiter ce sujet dans un texte Ces règles européennes peuvent être modifiées ou interprétées différemment à l'occasion d'actes de la Commission ou d'audits réalisés par la Commission. L'objectif du Gouvernement est bien de préciser pour la nouvelle PAC, qui commence en 2023, les conditions d'éligibilité des projets agrivoltaïques

Nous aurions aimé que la même attention soit portée à notre groupe et nous regrettons cette façon de faire, assez peu républicaine à notre sens. En tout état de cause, sur le fond, les sénateurs socialistes sont très attachés à ce que les aides de la PAC servent avant tout à accompagner les agriculteurs qui produisent des biens alimentaires. La situation économique difficile, voire parfois catastrophique, de nombreux agriculteurs français ne nous autorise clairement pas à détourner certaines aides européennes de leur nature première. À ce sujet, je tiens à rappeler que, lorsqu'il est question de la PAC et des aides du premier pilier, nous devons toujours raisonner en enveloppes fermées.

Il en va d'ailleurs de même lorsqu'il est question d'évaluation de nos politiques publiques- j'en prends pour témoin notre collègue Franck Montaugé, qui a déposé une proposition de loi constitutionnelle relative à ce sujet en 2021. C'est pourquoi, dans un souci de préservation de l'activité agricole, nous souhaiterions que tout soit mis en oeuvre afin d'éviter qu'une installation agrivoltaïque, une fois autorisée, ne fasse plus jamais l'objet de contrôles, ce qui ouvrirait la voie à des dérives certaines. Si nous ne pouvons pas aborder directement, dans le présent texte, la question des moyens financiers et humains pour y parvenir, nous demandons que le futur décret

La limitation à un mégawatt de l'éligibilité des installations agrivoltaïques à l'obligation d'achat, telle que proposée dans cet amendement, n'est pas souhaitable. En premier lieu, elle serait beaucoup plus restrictive plus restrictive que le droit existant, puisque les appels d'offres actuels de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en matière d'énergie solaire vont jusqu'à huit mégawatts. De plus, la commission n'a pas strictement fixé de seuils à un et six mégawatts pour l'agrivoltaïsme, mais a prévu un plafond et un décret : celui-ci pourra donc, en fonction des besoins des professionnels, fixer un seuil inférieur à ce plafond. Par ailleurs, le seuil de six mégawatts, issu des lignes

répond à une attente très forte de l'ensemble des acteurs de l'agrivoltaïsme, qui veulent favoriser le développement du secteur dans la durée et permettre un passage à l'échelle.

à la conversion à l'agriculture biologique des parcelles sur lesquelles sont implantés ces panneaux photovoltaïques. Il faut avant tout faire reculer l'usage des pesticides, qui- nous le savons -sont responsables d'une grande partie de l'effondrement de la biodiversité. Nous devons reconquérir

Un mécanisme de compensation est prévu par le code rural et de la pêche maritime. Il déclenche le mécanisme d'une étude préalable agricole qui suit les étapes suivantes : évaluation de la perte de potentiel financier agricole, estimation du délai nécessaire à sa reconstitution, calcul de l'investissement nécessaire à la compensation de cette perte. En tant que forme de photovoltaïsme, l'agrivoltaïsme doit logiquement être soumis à un tel mécanisme. Au demeurant, pour être qualifiée d'agrivoltaïque, une opération devra apporter la preuve

à des constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole, notion consacrée par le code de l'urbanisme et interprétée par la jurisprudence de manière à faciliter l'implantation du photovoltaïque sur les terrains agricoles. telle assimilation nous semble trop extensive : la production agricole doit rester la principale activité de l'exploitation, par rapport à la production d'énergie. Le présent amendement vise donc à supprimer les modifications apportées au code de l'urbanisme.

Le développement de l'agrivoltaïsme doit s'effectuer en concertation non seulement avec les agriculteurs, mais également- c'est très important ! -avec les collectivités, qui sont les garantes de l'acceptabilité sociale des projets. Les CDPENAF sont des institutions parfaitement adaptées pour favoriser le dialogue local. Il convient de les conforter dans ce rôle. On ne peut pas imposer aux agriculteurs et aux

n° 48 rectifié. Cet amendement a pour objet de permettre l'élaboration de chartes départementales relatives à la mise en oeuvre des projets agrivoltaïques.

donnera un avis sur le caractère nécessaire à l'exploitation agricole des installations agrivoltaïques.

Certaines d'entre elles présentent un profil qui devrait permettre d'installer de l'agrivoltaïsme. Cet amendement vise à prévoir une exception au principe de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante prévu

n° 14 rectifié. Le présent amendement a pour objet de soumettre tout projet d'installation agrivoltaïque à l'étude préalable en matière agricole prévue par l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.

Redon-Sarrazy. Cet amendement d'appel vise à demander la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur deux problématiques importantes qui ne peuvent pas être traitées au détour de la présente proposition de loi. La première est la nécessité d'anticiper au mieux les situations dans lesquelles un projet impliquerait plusieurs acteurs, à savoir un exploitant agricole, un propriétaire foncier agricole et un porteur de projet d'énergie solaire. Tout au long des débats, nous avons voulu mettre en avant la nécessité de préserver les agriculteurs et de ne pas détourner les terres agricoles de leur vocation première. En conséquence, aucun projet ne doit pouvoir être mené sans concertation ni accord de toutes les parties prenantes. De plus, il faut nécessairement que la répartition de la valeur ajoutée induite par la mise en place d'une installation photovoltaïque se répercute à la hauteur des efforts consentis par toutes les parties prenantes, plus particulièrement par l'exploitant agricole qui y sera confronté au quotidien. Actuellement, des chartes de bonnes pratiques existent pour réguler les relations et encourager la complémentarité entre agriculture et production photovoltaïque. Il faudrait en tirer un bilan et, en fonction de celui-ci, voir si elles ne peuvent pas être généralisées. La deuxième problématique que nous souhaitons aborder concerne les relations entre les communes et leurs groupements lors de l'émergence d'un projet sur un territoire. Nous souhaitons que tous les échelons, particulièrement les communes, soient toujours associés et informés au préalable. Par ailleurs, le sujet qui nous occupe aujourd'hui nous renvoie nécessairement à des questions financières, en particulier celle de la répartition de la fraction de la composante de l'Ifer. C'est un sujet central qui captera sans aucun doute l'attention sur le terrain. Il faudra nécessairement veiller à une juste répartition. Quel est

proposition de loi en faveur du développement de l'agrivoltaïsme, Mme

groupe GEST est constante : sobriété, efficacité et décarbonation par le biais des énergies renouvelables. L'agrivoltaïsme est un élément incontournable pour atteindre les objectifs de la PPE. Toutefois, nous entendons pleinement les inquiétudes de nombre d'agriculteurs,

Nous organisons demain au Sénat un colloque consacré à l'agrivoltaïsme. Nous espérons trouver de nouvelles mesures pour mieux encadrer son développement.

des avis défavorables. Néanmoins, dans la mesure où la proposition de loi garantit la protection des intérêts agricoles tout en permettant la production d'électricité par le développement d'un agrivoltaïsme respectueux de l'environnement,

Dans la discussion générale, la parole est Mme Vanina Paoli-Gagin, auteur de la proposition de loi. Monsieur

et à sortir des schémas habituels. Ce soir, nous devons travailler en conscience de l'urgence du long terme, pour reprendre l'expression d'Étienne Klein. La forêt doit s'adapter plus rapidement aux changements que le climat déréglé lui impose. Tant qu'elle évolue, elle est vivante. Sera-t-elle assez rapide pour lutter contre les maux qui l'attaquent ? Nous proposons, avec cette proposition de loi, d'amorcer une réflexion différente et d'apporter une première réponse, certes partielle, mais opérationnelle, à cet enjeu. Mes premiers remerciements vont à notre collègue Anne-Catherine Loisier, dont l'expertise et les conseils avisés ont fortement contribué au calage de ce texte. Je remercie aussi notre rapporteur et les membres de la commission des finances, dont je salue le vote très largement favorable à cette initiative. Nous sommes tous d'accord : la forêt apporte des bienfaits inestimables à notre environnement. Seules certaines de ses externalités positives sont visées dans l'exposé des motifs. Bien entendu, Bien entendu, j'ai pensé à la captation du carbone, à la contribution à la préservation de notre biodiversité ou encore à l'amélioration de la qualité de l'eau le filtrage naturel qu'assure la forêt.

Partant, agir efficacement pour accompagner la forêt devient une priorité pour notre pays. De ce chef, sa gestion durable est primordiale. Nous avons eu de nombreux échanges avec des acteurs clefs de la forêt et de ses filières amont et aval. Pour ma part, j'en ai également eu en ma qualité de présidente des communes forestières de l'Aube. Ce qui ressort de ces entretiens, c'est la complexité à embrasser et à traiter le sujet : c'est logique à l'aune des multifonctionnalités de la forêt. Ce texte est comme la première pierre de l'édifice qu'il nous faut bâtir ensemble : une première étape que nous avons choisi de cibler sur les forêts communales, parce que nous sommes ici, au Sénat, les représentants des territoires. tel fléchage était important à plusieurs égards. D'abord, parce que le manque de moyens de la plupart des communes rurales est un fait. parce que nous avons voulu notre dispositif incitatif en ce qu'il pose comme prérequis le régime forestier, assurant la sanctuarisation des forêts publiques et permettant une gestion planifiée. En outre, car je crois beaucoup à l'alliance public-privé dans des causes aussi justes que cet impératif de gestion durable. C'est important dans la société dans laquelle nous vivons et aspirons à nous définir. Enfin, parce que c'est, pensons-nous, une attente de nos concitoyens. Les événements récents, notamment les feux de forêt, qui ont ravagé près de 65 000 hectares cet été, ont suscité, à juste titre, de vives émotions. Les citoyens s'engagent, veulent participer à l'amélioration de leur environnement. Ils le prouvent en faisant des dons à des associations. Autant qu'ils puissent le faire, plus directement, auprès de leurs communes forestières, syndicats et groupements forestiers. Qu'ils le fassent en faveur de leur forêt de résidence ou de coeur, contribuant ainsi au financement du rachat de parcelles, de replantations, d'aménagements d'accès, etc. Les maires et acteurs auditionnés ont montré leur enthousiasme pour les mécanismes de dons par des personnes physiques et morales proposés aux articles 1 et 2 du texte. Certains nous ont confié qu'ils attendaient, de longue date, un tel dispositif. Preuve en est, s'il le fallait, de l'utilité de notre démarche. Nous apportons un supplément de clarté juridique, afin de lever tout flou et de permettre une pleine application de la loi au bénéfice des forêts communales.

Chacun doit se sentir concerné et disposer de moyens d'action. C'est en tout cas la vision que nous partageons au sein du groupe Les Indépendants. Nous pensons l'écologie libérale, où les forces en présence dégagent des solutions de progrès, n'opposant pas environnement, société et économie. Nous souhaitons, par notre approche holistique, tracer le chemin d'un possible pour les générations suivantes. Pour contribuer à cet équilibre de la forêt, nous vous invitons, mes chers collègues, à participer à l'examen des articles du texte

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il nous revient ce soir d'examiner la proposition de loi de notre collègue Vanina Paoli-Gagin visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt.

avec son auteur. Il devait en être ainsi, car cette proposition de loi s'inscrit dans un contexte lourd, que nous connaissons tous : l'augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes et des incendies qui y sont associés, ainsi que la crise sanitaire due aux scolytes. Si cette gestion durable ne constitue pas la garantie d'une défense absolue contre tous les dangers qui assaillent une forêt, par définition vulnérable, elle permet de les contenir. Havre de biodiversité et puits de carbone, la forêt constitue un bien qui n'est pas estimé à sa juste valeur par le marché. La proposition de loi vise ainsi à mieux valoriser certaines de ses externalités positives en incitant, par une réduction d'impôt, les particuliers et les entreprises à donner aux communes et syndicats forestiers pour financer certaines des opérations de gestion Elle concerne donc à la fois une part importante de la forêt française, les forêts communales représentant près de 15 % de la surface forestière de France métropolitaine, et une part modeste, puisqu'elle ne permet pas de soutenir la gestion de la forêt guyanaise, vaste de 8,3 millions d'hectares, mais principalement domaniale, donc relevant de l'État. Nul doute toutefois que la présente proposition de loi va dans le bon sens et apporte une pierre nécessaire à l'édifice. L'ensemble des questions soulevées par la gestion de la forêt nécessiterait sans doute à l'avenir une grande loi sur Mais si l'on peut, en attendant, pousser les particuliers et les entreprises à réaffirmer par le mécénat le lien qu'ils entretiennent avec leur commune et avec leur forêt, on aura fait oeuvre utile. C'est le sens de la proposition de loi. Avant d'entrer dans l'examen du texte, j'aimerais rappeler brièvement comment sont gérées les forêts communales et comment est financée cette gestion. Les forêts communales représentent 2,8 millions d'hectares sur les 17 millions que constitue la forêt métropolitaine sont gérées, lorsque la loi est bien appliquée, dans le cadre du régime forestier. Celui-ci définit les grandes règles qui visent à assurer la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine. Sa mise en oeuvre est confiée à un opérateur unique, l'Office national des forêts (ONF), qui est chargé de garantir une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt : économique, par la vente de bois ; écologique, notamment par la préservation de la biodiversité ; sociale, par l'accueil du public. Ce régime repose sur un financement commun des communes et de l'État. D'une part, les communes versent à l'ONF des frais de garderie, ainsi qu'une contribution annuelle de 2 euros par hectare de terrain relevant du régime forestier. D'autre part, l'État octroie un versement compensateur, qui vise à couvrir la différence entre le coût pour l'ONF et les contributions le coût pour l'ONF et les contributions des communes. Le surcoût des actions d'aménagement excédant celles qui sont prévues par le régime forestier est assumé par les communes sur leurs ressources propres, avec le soutien éventuel d'autres collectivités ou de l'État. Si certaines communes parviennent à se ménager des recettes substantielles, qui vont de pair avec des essences productrices et une culture forestière historique- on peut ici penser aux communes des Landes -, il faut avoir en tête que la gestion d'une forêt n'est pas toujours rentable, tant

Elle a entraîné une chute des recettes forestières des communes au moment où elles en ont le plus besoin. On comprend alors que les Assises de la forêt et du bois aient mis en évidence, au mois de mars dernier, le besoin de financements supplémentaires. Cette Cette proposition de loi arrive ainsi à point nommé. Elle vise à appliquer la réduction d'impôt au titre du mécénat des particuliers et des entreprises aux dons versés aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers, forestiers, pour l'entretien, la reconstitution ou le renouvellement des bois et forêts présentant des garanties de gestion durable. Seraient également éligibles à la réduction d'impôt les dons venant financer l'acquisition des parcelles dont la gestion n'est pas nécessairement durable, mais a vocation à le devenir. Cela permettrait aux communes d'acquérir des forêts parfois laissées à l'abandon. Par anticipation sur la discussion des amendements, je rappelle ici que l'entretien des forêts participe à la prévention et, finalement, à la lutte contre les incendies. Si le dispositif prévu par cette proposition de loi paraît en partie satisfait, il est, dans les faits, peu utilisé. Il est peu ou pas connu des particuliers et des entreprises, qui préfèrent donner à des fonds de dotation bénéficiant d'une meilleure visibilité. De même, les communes forestières qui disposent de peu de moyens juridiques ne sont probablement pas en état de saisir que les opérations de gestion forestière qu'elles mènent sont susceptibles d'être financées par des dons éligibles à une réduction d'impôt. La mise sur pied d'un système de financement pouvant s'appuyer sur ces dons serait d'ailleurs lourde et incertaine. Supposant le recours au rescrit fiscal, elle dépendrait alors de l'interprétation casuistique de l'administration fiscale.

loi s'attache simplement à soutenir l'action des communes forestières, qui, pour certaines d'entre elles, peuvent se trouver financièrement en difficulté à l'heure où la gestion durable de la forêt constitue un défi sans précédent. Le coeur du financement de cette compétence doit demeurer une combinaison entre les contributions de la commune et le versement compensateur de l'État. En revanche, si les particuliers et les entreprises peuvent « mettre la main à la pâte » et contribuer davantage à la bonne gestion de la forêt, s'ils peuvent ainsi, modestement, ici éviter un ici éviter un incendie, là ralentir la propagation d'un parasite, il faut l'encourager. Cette proposition de loi n'est pas le « grand soir » de la forêt, mais, je le répète, si l'on peut pousser les particuliers et les entreprises à réaffirmer par le mécénat le lien qu'ils entretiennent avec leur commune et avec leur forêt, on aura fait oeuvre utile.

ou encore à la crise sanitaire due aux scolytes, mettent en lumière les défis importants qu'il nous faut relever pour mieux gérer et préserver ce bien unique qu'est notre forêt. Unique, parce qu'il s'agit non seulement d'un élément constitutif de notre patrimoine, mais aussi parce que la forêt, comme le soulignent les auteurs de la proposition de loi, est porteuse d'externalités positives. Je pense en premier lieu à la captation de carbone, qui constitue un atout extraordinaire pour accélérer la transition écologique et lutter contre le changement climatique. Je pense également à la préservation ou à la restauration de notre biodiversité que permettent nos forêts et leurs sols. Je pense aussi, et c'est un aspect sans doute moins évoqué,

s'inscrit dans cet esprit. Vous en préconisez de renforcer les capacités financières des collectivités propriétaires de forêts, qui représentent 10 % de la forêt française, afin de les aider à répondre à ces défis, par la mobilisation de dons. Je voudrais le dire de la manière la plus claire qui soit : il ne s'agit ni dans notre esprit ni dans le vôtre de substituer des financements privés à des financements publics, qui demeurent nécessaires. Il nous semble au contraire que les deux sont complémentaires, comme M. le rapporteur vient de le dire. Nous saluons l'idée de financements de proximité, par des citoyens ou des entreprises qui reconnaissent les externalités positives de leur territoire. C'est bien l'enjeu de ce texte.

de la sénatrice Vanina Paoli-Gagin et du rapporteur Vincent Segouin. Je tiens également à souligner le lien qui est fait, à l'issue des travaux de la commission, avec les documents de gestion durable durable prévus par le code forestier. Il s'agit effectivement de la pierre angulaire de la politique forestière nationale, dans le contexte du changement climatique et pour faire face au risque grandissant des incendies. Je sais le Sénat particulièrement mobilisé sur cette question. La rédaction choisie permet de répondre avec cohérence aux attentes légitimes de garantie d'une gestion durable et multifonctionnelle. Par ailleurs, la condition est remplie pour les forêts publiques relevant déjà du régime forestier et d'une gestion par l'ONF. Il faut qu'elle le soit pour les forêts publiques, qui devraient relever du régime forestier et qui n'y sont pas encore. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement accueille votre proposition de loi avec bienveillance et s'en remettra à la sagesse du Sénat. Je tiens enfin à insister devant vous sur l'engagement du Président de la République et de la Première ministre. Je pense au déploiement des Assises de la forêt et du bois, qui qui doit être notre perspective, mais aussi au grand chantier national de la reconstruction d'un certain nombre de forêts détruites par les incendies, qui va débuter. Nous avons un intérêt collectif à expliquer ce que signifie gérer durablement la forêt et les sols forestiers. La forêt est un trésor à bien des égards : biomasse, ressources, biodiversité, services écosystémiques,

sécheresse après sécheresse, attaque après attaque. Les mesures de renouvellement forestier de France Relance et, à présent, de France 2030 visent à accompagner ces transitions sur le long terme et de façon pérenne. Il faut enfin l'adosser à des filières résilientes, compétitives et rentables. Le secteur devra faire face à plusieurs enjeux : évoluer et s'adapter à la nouvelle donne des marchés, notamment de l'énergie, dans une vision de long terme, afin de contribuer à la décarbonation de notre économie. Il doit gagner en agilité dans son adaptation aux conditions du marché et de la demande, intégrer les fluctuations de récoltes liées aux impacts des aléas, comme les tempêtes, les incendies, les dépérissements, et adapter les essences aux besoins des massifs forestiers français. développer enfin ses capacités de transformation et de production de produits plus innovants pour lesquels la demande existe, au regard des tendances de marché, et à plus forte valeur ajoutée, pour décarboner notre économie, notamment dans la construction. dans la construction. La planification est indispensable pour repenser l'écosystème forestier et fonder une politique forestière efficace. C'est d'autant plus fondamental dans ce contexte de rapide transformation et de changement climatique, où la plupart de nos référentiels techniques sont remis en cause. Je vous remercie de cette proposition de loi, qui permet de tracer un chemin sur l'un des volets de la politique forestière.

monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le texte présenté par notre collègue Vanina Paoli-Gagin dans un contexte où les conséquences du changement climatique sur la gestion des forêts sont de plus en plus perceptibles par l'opinion publique. Je ne reviendrai pas sur les feux de forêt qui ont rythmé les actualités de notre pays tout au long de la période estivale, mais il est important de noter que nous sommes, sans mauvais jeu de mots, dans une actualité brûlante en la matière. Des Cévennes aux Bouches-du-Rhône en passant par la Gironde, des feux importants, considérés par la communauté scientifique comme des « mégafeux », ont détruit plus de 11 000 hectares de forêt cet été. À l'échelon mondial, les prévisions de l'ONU, comme celles du Groupe d'experts Ces incendies ont des conséquences importantes, dans la mesure où ils entraînent la disparition de plusieurs espèces animales et végétales. L'exemple australien est révélateur : les « mégafeux » de brousse de 2020 auraient causé la disparition de milliards d'animaux ainsi que de 832 espèces différentes. Cette proposition de loi, qui a trait au régime des dons octroyés à des communes ou établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de la gestion de la forêt, s'insère donc dans un moment décisif. Elle vise ainsi, par un accroissement des dons, à mieux financer l'entretien de la forêt publique, qui représente- rappelons-le -seulement un quart environ de la forêt française. Plusieurs remarques me viennent à la lecture du texte. Tout d'abord, le ciblage nous paraît très largement imparfait par rapport à l'ambition développée dans l'intitulé et dans l'exposé des motifs. Ensuite, le texte vise à faire supporter le financement de l'action publique par les dons, et non par la puissance publique. Je reviendrai plus longuement par la suite sur les raisons qui me poussent à penser que cela n'est pas la bonne doctrine.

de loi intervient à un moment où la forêt française est à la croisée des chemins, comme l'a été l'agriculture dans les années 1950. Nous allons devoir collectivement prendre des décisions. Dans les décisions. Dans les années à venir, il va falloir choisir entre un modèle industriel d'exploitation et un modèle pérenne de sylviculture douce qui respecte la multifonctionnalité des forêts. Alors que nous n'avons de cesse de parler de décarbonation de notre économie afin de baisser nos émissions de CO2, il n'est pas inutile de rappeler que les arbres séquestrent et stockent du carbone grâce à la photosynthèse, et libèrent en retour de l'oxygène. En un an, un arbre peut absorber entre 10 et 20 kilogrammes de CO2. CO2. Au-delà de la fonction écologique, c'est aussi la fonction sociale de la forêt qui doit être mise en exergue, car nos forêts accueillent chaque année près de 700 millions de visites. Pour protéger ces vecteurs sociaux et écologiques, il faut un État fort et présent. Or la situation de l'ONF est plutôt révélatrice du désengagement de l'État en la matière. En vingt ans, cet organisme a connu près de 5 000 suppressions de postes. Et il semble que le mouvement soit bien parti pour durer, le Gouvernement ayant décidé l'an dernier de supprimer 500 emplois supplémentaires sur cinq ans.

car le dérèglement climatique et le dépérissement des forêts vont nécessiter de plus en plus de travail, comme le suivi sanitaire et le renouvellement des peuplements forestiers. Derrière ces suppressions de postes se cache aussi un malaise bien plus profond et dramatique chez ceux qui, par leur passion, entretiennent et protègent nos forêts. Entre 2005 et 2020, cinquante et un agents de l'ONF ont mis fin à leurs jours. Ce taux est deux fois plus élevé que dans le reste de la population française. Le malaise est révélateur de l'état de la profession. Les suicides ne peuvent pas s'expliquer par la seule solitude du forestier isolé dans les bois. La profession a le sentiment que la mutation dont elle fait l'objet l'aliène. de la sémantique est éloquente : le terme de « garde forestier » a été remplacé par celui d'« agent patrimonial ». À la base, les gardes forestiers étaient là pour garder la forêt, afin de tout gérer de manière généraliste sur un territoire donné. Désormais, l'agent patrimonial est spécialisé sur le terrain, divisé, branche par branche, et soumis à l'objectif permanent de rendement. C'est précisément cela qui crée une perte d'identité significative. C'est donc cette logique comptable, poussant au demeurant éternellement aux rendements toujours plus considérables et à la financiarisation de l'exploitation forestière, qui est permise par une ouverture toujours plus grande aux entités privées dans ce domaine pourtant commun. Pour conclure, bien que le sujet, ainsi que le principe qui le sous-tend semblent bons, je déplore le manque d'ambition de la proposition de loi, dans la mesure où le texte se cantonne à une part réduite de la forêt française et ne retient pour seul mécanisme que la réduction fiscale. Réduction qui s'inscrit dans un contexte où le Gouvernement organise perpétuellement l'attrition des finances publiques. Le désarmement fiscal ne saurait être une réponse satisfaisante aux limites de financement des politiques publiques,

La déforestation est à l'oeuvre en France, même si le patrimoine forestier est davantage préservé qu'ailleurs sur la planète. Il a été préservé, entre 1990 et 2020, par la régénération naturelle. Mais l'intervention humaine est défaillante dans la sauvegarde de nos forêts, qu'elles soient en plantation ou plus anciennes.

entre 2010 et 2019. La situation est paradoxale. Dans son dernier rapport annuel, le Haut Conseil pour le climat relève que « la dégradation significative de la capacité des forêts à capter du carbone a réduit les absorptions de CO2 de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) à leur niveau de 1990 ». En 2017, la capacité d'absorption des puits de carbone s'est effondrée entre 3 % et 4 %, soit trois fois moins qu'en 2005. On recule à une telle allure que l'objectif de 9 % en 2020 est caduc, et celui de 13 % en 2030 est hors d'atteinte. Le législateur est dès lors bien fondé à intervenir pour enrayer ce phénomène annonciateur d'un désastre climatique. La proposition de loi que vous nous soumettez entendait, avant son passage en commission, se focaliser sur les communes forestières, soit à 15 % des hectares forestiers. rien dans ce texte sur les forêts domaniales ni, plus grave, sur les forêts privées, qui représentent les trois quarts du domaine forestier français. Nous voterons contre ce texte, qui s'inscrit dans la plus stricte idéologie néolibérale, sans aucune solution nouvelle. L'exposé des motifs a le mérite d'être clair : « En la matière, l'État ne peut pas tout. Cette proposition de loi répond d'une écologie libérale de progrès, basée sur les innovations et la recherche, ainsi que sur une implication collaborative des secteurs public et privé. » Sans surprise, Sans surprise, le texte se borne à envisager deux dispositifs de mécénat, l'un pour les particuliers, l'autre pour les entreprises, le tout payé par le contribuable les réductions d'impôt prévues. Franchement, pensez-vous qu'il soit possible de sauver les communes forestières en grignotant les recettes de l'État ? Nous ne devrions pas avoir à choisir entre les coupes rases forestières et les coupes rases de nos finances publiques. Vous créez une niche fiscale de plus. Il en existait déjà 180 ; en voilà une nouvelle ! Peut-être l'ignoriez-vous, mais votre dispositif existe déjà les communes peuvent déjà recevoir des dons des particuliers et des entreprises dans les conditions que vous prévoyez. Le donateur, c'est d'ailleurs une condition, indique que son don doit être strictement affecté à l'objet souhaité. En l'occurrence, ici, ce serait le renouvellement et l'entretien des forêts. J'ai vérifié, c'est une mesure sans contrôle fiscal et

peu de raisons de croire à un ruissellement nouveau pour les forêts. Je crois que les fondements idéologiques sur lesquels repose ce texte sont incompatibles avec l'ambition affichée. même récit, où les agents économiques seraient mieux à même que la puissance publique de décider ce dont la société a besoin. Il conviendrait pour eux d'arbitrer entre différentes causes. En somme, le capital choisirait ses engagements. Des gestes librement consentis constitueraient une alternative vertueuse à l'impôt tant décrié, pour mener les défis qui se posent à la biodiversité et au patrimoine forestier. La contribution serait volontaire, au lieu d'être une collecte subie. Croyez-vous vraiment que les communes forestières manquent de moyens parce qu'elles manquent de dons privés ? ? Non ! Les communes forestières pâtissent, comme les autres, peut-être plus encore, de la baisse des concours financiers de l'État par la DGF. Cette baisse, monsieur le ministre, a été de 23,4 % en moyenne sur la période 2013-2017, mais

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la dernière loi d'orientation sur la forêt remonte à 2001, bien que je n'oublie pas la prise en compte de tels enjeux dans les grandes lois agricoles ou environnementales adoptées depuis. Cependant, au regard de certaines difficultés structurelles persistantes et des terribles incendies de cet été, il est urgent d'y consacrer du temps, pour ne pas dire de l'argent. Aujourd'hui, il s'agit avant tout de contribuer à la préservation des externalités positives puits de carbone, sanctuaire de la biodiversité et refuge d'une eau à la qualité préservée ... Les nombreux atouts de la forêt nous imposent des devoirs. La gestion durable de la forêt est, bien entendu, le premier d'entre eux, sans quoi c'est-à-dire son exploitation économique ou son usage social, seraient irrémédiablement hypothéqués. La proposition de loi va dans ce sens, à travers l'incitation fiscale. Mon groupe est favorable à tout ce qui pourrait encourager le mécénat des particuliers et des entreprises, sous réserve que cela ne conduise pas l'État à se désengager de ses propres responsabilités. La forêt, bien qu'elle se divise entre statut domanial, public ou privé, est un bien commun. L'action publique doit donc veiller à la cohésion de sa gestion sur l'ensemble du territoire, avec, d'un côté, des moyens financiers à la hauteur des enjeux, et, de l'autre, les bonnes réponses à ses handicaps, dont le problème du morcellement ; j'y reviendrai. question du financement. Le régime forestier est-il suffisant à soutenir toutes les opérations nécessaires à la gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques ? Visiblement non, puisqu'il faut faire appel aux dons. Nous constatons en effet qu'une partie des communes forestières ont des dépenses supérieures aux recettes.

Les contrats d'objectifs incitent aux regroupements, mais nous sommes loin d'avancer sur ce terrain. Il faudrait promouvoir davantage les instruments existants tels que les groupements forestiers, les organismes de gestion en commun ou encore les organisations syndicales.

Monsieur le ministre, votre prédécesseur avait lancé les Assises de la forêt et du bois afin de « construire une vision ambitieuse et partagée pour la forêt française de 2030 ». J'espère que des propositions seront rapidement sur la table. En attendant, le groupe RDSE votera cette proposition de loi. Très

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nos forêts sont une composante à part entière de nos paysages et de notre patrimoine national. Elles couvrent 31 % de notre territoire, soit 17 millions d'hectares en métropole, et 8,7 millions d'hectares en outre-mer. Elles abritent évidemment une incroyable biodiversité, mais sont aussi de véritables puits de carbone, captant et stockant au moins 12 % des émissions de gaz à effet de serre en France La France a su instaurer très tôt une gestion durable et équilibrée de la forêt, en favorisant le développement d'une filière bois compétitive et créatrice d'emplois. Nous disposons ainsi d'une production nationale en bois à l'heure où les prix sur le marché ne cessent de grimper. Mais ces espaces, si indispensables pour notre pays, ont été extrêmement fragilisés par le réchauffement climatique. Les forêts du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté sont particulièrement touchées par le scolyte, un insecte qui creuse sous l'écorce de l'arbre jusqu'à le tuer. Au total, 50 000 hectares ont officiellement périclité depuis 2018, et d'autres régions sont également touchées en raison des sécheresses. L'autre effet, plus visible, du réchauffement climatique, ce sont les incendies. L'année 2022 a été particulièrement marquée par des épisodes de sécheresse ayant entraîné d'importants feux de forêt.

la surface brûlée pourrait ainsi augmenter de 80 % d'ici à 2050. En France, 15 % des forêts sont gérées par des collectivités locales, ce qui représente 14 000 forêts communales pour une surface de 2,8 millions d'hectares. Les dépenses du bloc communal pour l'entretien des forêts s'élèvent à environ 110 millions d'euros en 2021. En raison des incendies et du scolyte, les recettes des communes forestières sont en nette diminution. Elles sont passées de 178 millions d'euros en 2019 à 153 millions d'euros en 2020, conduisant 30 communes à enregistrer en 2021 une épargne nette négative. Certaines forêts communales, notamment dans le sud de la France, nécessitent d'importantes dépenses pour la défense contre les incendies. Près de 35 millions d'euros sont ainsi financés chaque année par les départements et les communes. La proposition de loi que nous examinons intervient dans ce contexte et vise à renforcer la faculté des personnes physiques et morales à participer à la gestion durable des forêts gérées par les collectivités. La commission des affaires économiques, dont je salue le travail, a conservé et renforcé les articles 1 et 2, visant à appliquer la réduction d'impôt au titre du mécénat des particuliers et des entreprises aux dons versés aux communes et syndicats intercommunaux de gestion forestière,

La commission des affaires économiques a d'ailleurs choisi d'élargir le dispositif présenté dans la proposition de loi en étendant la réduction d'impôt aux dons versés aux syndicats mixtes et groupements syndicaux forestiers, ces derniers pouvant respectivement comprendre une commune ou avoir été constitués avec l'accord d'une commune.

Les dispositions qui permettront de renforcer la participation de nos concitoyens et de nos entreprises à leur gestion et au soutien des collectivités ne peuvent qu'être saluées. C'est pourquoi je voterai cette proposition de loi. Excellent